ans maire de Carnac- tout un symbole de solidité bretonne ! Élu à huit reprises député du Morbihan,

Au cours de ses deux mandats sénatoriaux, il fut une véritable référence au sein de la commission des lois. Il y fut le rapporteur incontournable de tous les textes concernant les questions électorales- sujet d'actualité

Mme la ministre du travail. Madame la ministre, depuis le début de la crise sanitaire, les personnels de santé, les caissiers, les livreurs, les éboueurs, les agriculteurs, les postiers et tant d'autres exposent chaque jour leur santé pour assurer les fonctions vitales du pays. Alors que leur sécurité sanitaire est loin d'être toujours assurée, vous appelez à la reprise de l'activité non essentielle. Mais avec quelles garanties sanitaires ? Les masques sont-ils arrivés en quantité suffisante ? Les entreprises sont-elles prêtes à s'organiser face à un risque biologique invisible ? Quel accompagnement l'État Repenser l'organisation du travail, comme la justice l'a rappelé à Amazon, est une nécessité impérative. Dans ce contexte, l'inspection du travail est indispensable pour accompagner les entreprises et garantir la sécurité sanitaire des travailleurs. Pourtant, au lieu de donner aux inspecteurs les moyens d'exercer leurs missions, vous entravez honteusement leur action. En effet, la direction générale du travail (DGT) exige désormais des inspecteurs qu'ils fassent valider par leur hiérarchie toute visite en entreprise ou toute saisine du juge des référés, une disposition contraire à la convention n° 81 de l'Organisation internationale ressources humaines de votre ministère a suspendu l'inspecteur Anthony Smith. Sa « faute » ? Exiger d'une entreprise d'aide à domicile, après une alerte des représentants du personnel, qu'elle fournisse des masques pour protéger salariés comme usagers- Ces pressions inacceptables font l'objet d'une plainte- légitime -contre la France transmise par quatre syndicats au Bureau international du travail. Madame la ministre, nous vous demandons d'abroger les ordres illégaux de la DGT, d'abandonner les sanctions et menaces qui pèsent sur les inspecteurs du travail et de leur fournir les moyens juridiques et matériels de travailler en sécurité. Ce sont des prérequis impératifs à la reprise

Le 17 mars, la direction générale du travail, qui est l'autorité centrale de l'inspection du travail conformément aux règles de l'OIT, a donné des instructions pour assurer

les salariés et conseiller les entreprises. C'est bien dans ce cadre que l'inspection du travail fonctionne. Vous m'interrogez aussi sur un cas particulier. La direction générale du travail a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire un inspecteur du travail de la Marne, qui avait enfreint à plusieurs reprises et de façon délibérée et grave les instructions de l'autorité centrale. Il avait enjoint à des employeurs des conditions de maintien d'activité contraires aux prescriptions des autorités sanitaires, il était intervenu hors de sa compétence et il avait eu des pratiques internes non déontologiques par rapport aux instructions.

La culture est en danger. Beaucoup de ses artistes, intermittents, techniciens et auteurs ainsi que les structures qui les emploient sont déjà en mode survie. Pourtant, culture ne s'est jamais révélée aussi essentielle que dans cette période de confinement : au travers de leurs créations numériques et grâce à la qualité de notre audiovisuel public, les créateurs nous enchantent quotidiennement et nous aident à résister. Mais l'été sera sûrement silencieux et l'automne s'annonce très périlleux, car incertain.

qu'est-ce qu'un « petit » festival ? -pourraient avoir lieu après le 11 mai que vous rassurez les acteurs, les organisateurs, mais aussi les collectivités territoriales, lesquelles sont depuis le début en première ligne et ne demandent qu'à être associées.

ne peut attendre vous avez raison : le secteur de la culture est particulièrement touché par cette crise. C'est évidemment dramatique, d'un point de vue tant économique et social que sociétal et psychologique. Je pense à tous les artistes et à toutes celles et tous ceux qui travaillent dans le secteur culturel, qui voient

Depuis le début de cette crise, le ministère de la culture, en liaison avec les autres ministères et sous l'autorité du Premier ministre, a fait en sorte que tous les dispositifs transversaux puissent accompagner les secteurs de la culture. Nous avons veillé à ce que les intermittents, les auteurs, tous les acteurs de la culture bénéficient d'une manière ou d'une autre de ces dispositifs.

nous aurons besoin de continuer à travailler ensemble, Gouvernement, collectivités territoriales, acteurs de la culture, parlementaires ... Nous devons réussir ensemble ce rebond

madame Robert,

faisons attention, monsieur le ministre ! La parole est à M. Jérôme Bignon, pour le groupe Les Indépendants-République et Territoires. alors que le confinement semble produire ses premiers effets et autorise un optimisme prudent, les professionnels de santé s'alarment de la désertification de leurs cabinets. maladie (CNAM) a observé un recul de 40 % à 50 % de la consommation de soins, aussi bien en médecine générale que dans différentes spécialités. Vous l'avez vous-même souligné récemment. La filière cancérologie est particulièrement touchée. Dans la Somme, aucun dépistage de cancer du sein n'a été réalisé depuis le début du confinement. De nombreux patients renoncent à se rendre aux urgences par peur de la contagion.

De nombreux praticiens appellent à une réévaluation de l'urgence des soins déprogrammés La rupture dans la continuité des soins est particulièrement dommageable pour les personnes âgées et/ou handicapées. Faute d'équipements de protection suffisants, les aides à domicile n'assurent plus les soins courants pour ces personnes. Dans les maternités, le dépistage néonatal réalisé au troisième jour après la naissance- il permet une prise en charge précoce de cinq maladies graves désorganisé faute de portage postal efficace. Des retards de vaccination sont aussi observés chez les nourrissons et les jeunes enfants. Monsieur le ministre, une nouvelle vague de mortalité, différente, pourrait se dessiner. Pourriez-vous dresser

essentiels. Certains sont atteints de maladies chroniques ; d'autres ne sont pas malades, mais renoncent à des dépistages de cancers- cancer du sein, cancer colorectal. Des femmes enceintes n'ont pas forcément eu toutes les échographies obstétricales, dont elles doivent pourtant bénéficier.

que l'ensemble de la représentation nationale réaffirme, une fois de plus, son soutien à nos forces de sécurité. Dans cette crise sanitaire,

les règles du confinement doivent s'appliquer et être contrôlées de la même façon partout sur notre territoire, il n'y a pas de quartier dans lequel nos forces de sécurité intérieure n'interviendraient pas.

qui sont en cause au travers de ma question, mais le système. Comment expliquer que, deux mois après les expérimentations du professeur Raoult sur la chloroquine, on ne sache toujours rien sur l'efficacité de ce traitement, alors qu'une expérimentation massive aurait sans doute apporté des réponses depuis un mois ? Comment expliquer qu'il a fallu attendre un mois avant de répondre aux propositions des laboratoires vétérinaires pour tester plus largement les porteurs du Covid-19 ? Quinze jours après la levée des barrières administratives, leurs capacités ne sont toujours pas utilisées.

Tous ces dysfonctionnements sont liés à la gestion bureaucratique d'une administration qui croule sous les lois, les règlements, les protocoles, lesquels sont complètement inadaptés à une gestion de crise. Monsieur le ministre, gérer une crise, c'est oublier les contraintes administratives. Que comptez-vous faire pour accélérer le fonctionnement de notre système administratif et médical, aujourd'hui dépassé ? La parole est à M. le ministre des solidarités et de la santé.

Au moment où une crise sanitaire inédite frappe notre pays, entraînant ainsi le confinement de la population, nos pensées vont tout particulièrement aux plus vulnérables : nos enfants. Les chiffres, nous les connaissons : 130 000 filles et 35 000 garçons subissent des viols ou des tentatives de viols chaque année, en majorité incestueux 140 000 enfants sont exposés à des violences conjugales. Ces violences, elles ne s'arrêtent pas subitement durant le confinement. Au contraire, les risques sont décuplés par l'impossibilité pour l'enfant de trouver refuge durant la journée : à l'école, au sport ou chez des camarades de classe. Ces rares moments de répit, où l'enfant peut parler et échapper, ne serait-ce qu'un instant, aux violences qu'il subit, s'effacent, laissant place à la solitude la plus totale. Je pense également à ces milliers d'enfants suivis dans le cadre d'une action éducative en milieu ouvert et qui se retrouvent aujourd'hui vingt-quatre heures sur vingt-quatre avec leurs parents, malgré les tensions qui peuvent exister au sein des familles. Je pense aux travailleurs sociaux, qui, malgré leur dévouement le plus total, peinent à assurer leurs missions dans un contexte de crise sanitaire qui bouleverse nos modes de déplacement, et qui subissent depuis trop longtemps les coupes budgétaires dans un grand nombre de départements ces mêmes départements qui, de manière unilatérale et contre l'avis du juge, n'assurent plus les visites médiatisées et qui rompent totalement les liens entre les parents et les enfants depuis près d'un mois et demi ; ces mêmes départements qui, au début du confinement, ont renvoyé certains enfants dans leur famille malgré les risques encourus. Je vous le dis, car cette situation dramatique s'observe chez moi, dans les Hauts-de-Seine. Je pense enfin à ces milliers de jeunes isolés, hébergés dans des hôtels sociaux et dont les moyens matériels insuffisants ne permettent pas de suivre leurs enseignements au même titre que les autres jeunes. Face à cette situation, le Gouvernement, les associations et la société dans son ensemble se mobilisent. Monsieur le secrétaire d'État, vous avez multiplié les canaux permettant une meilleure détection des violences : je pense à l'adaptation du 119, permettant ainsi les signalements en ligne, à l'augmentation du nombre d'écoutants, grâce notamment au soutien des associations, et à l'élargissement du 114 pour les violences intrafamiliales. À cela vient s'ajouter la mobilisation des associations, des organisations non gouvernementales (ONG) et des collectifs d'anciens enfants placés qui luttent contre les violences et soutiennent les enfants en danger.

dernière. La famille, qui est ce lieu de protection, d'amour et d'épanouissement pour l'enfant, est aussi un lieu de maltraitance, de violences. Une augmentation de 89 %, cela ne nous surprend pas. C'est le signe de l'augmentation des violences pendant cette période de confinement, mais je veux y voir aussi le baromètre de notre vigilance accrue pour chacun d'entre nous. Deux autres chiffres vont dans ce sens. En effet, la semaine dernière, le nombre d'appels passés par les voisins a augmenté de 84 le nombre d'appels passés par des camarades a doublé, soit une augmentation de 100 %. Le formulaire en ligne que nous avons mis en place sur allo119.gouv.fr recueille chaque semaine plus de 200 saisines. Tout cela fonctionne, y compris les campagnes de communication que nous avons lancées auprès des Français ; mais encore faut-il que ces appels ne restent pas sans réponse.

Comme l'a très justement rappelé le Président de la République, et vous-même l'avez souligné, monsieur le Premier ministre, les collectivités locales représentent un maillon essentiel dans le dispositif de mise en oeuvre des mesures nationales et d'accompagnement des populations face à la crise du coronavirus. sociaux ou les centres communaux d'action sociale (CCAS) ont fait preuve d'une très grande réactivité dans des domaines comme le soutien aux familles en difficulté, le lien avec les populations fragiles, la livraison de repas à domicile ou de courses de produits de première nécessité, le contact régulier avec les personnes âgées ou isolées, ou encore l'acquisition et la distribution de masques. Les régions, en plus de leur participation au fonds de solidarité, ont pour la plupart mis en place des dispositifs complémentaires d'aides aux entreprises avec parfois des possibilités de délégation par convention aux départements, aux EPCI ou aux communes, comme dans les Hauts-de France. Cependant, beaucoup de petites structures, malgré leur éligibilité au fonds de solidarité, qui est indispensable, mais peut-être pas suffisant, seront confrontées pendant plusieurs mois à des difficultés récurrentes mettant en cause leur pérennité. Les interlocuteurs les mieux placés pour accompagner sur le plan économique ces microentreprises, autoentrepreneurs, travailleurs indépendants, artisans ou commerçants, seuls ou avec un ou deux salariés, semblent être les collectivités de proximité, c'est-à-dire les départements, les EPCI et les communes, qui peuvent le mieux appréhender leurs besoins. Toutefois, la législation ne leur permet pas aujourd'hui d'intervenir directement en soutien financier à ces petites entreprises sous la forme, par exemple, d'avances remboursables ou de prise en charge de loyers. Peut-on envisager, avec bien sûr un encadrement législatif et réglementaire strict, d'assouplir, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, les textes qui régissent l'exercice de cette compétence économique d'aide directe aux très petites

je vous remercie d'abord d'avoir rappelé le rôle important des collectivités territoriales. Vous m'interrogez plus précisément sur la participation financière aux entreprises des territoires. Comme vous le savez, c'est la région qui est compétente pour définir les aides, les régimes qui leur sont applicables, et pour attribuer les aides directes aux entreprises. Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent adopter des dispositifs d'aide immobilière aux entreprises, il faut aussi le rappeler. Par ailleurs, les EPCI

Les départements, en revanche, ne peuvent pas financer des aides aux entreprises, ni en mettant en place un fonds personnel ni en participant au fonds régional, sauf si ce fonds vise à financer les secteurs qui relèvent de la compétence du département- je pense par exemple à l'économie sociale et solidaire. Cette règle, il faut nous y tenir. En effet, dans cette période compliquée, nous ne devons pas disperser nos forces. Vous avez d'ailleurs rappelé vous-même le rôle très important des départements dans l'exercice des compétences sociales,

toutes les politiques sociales du département. Par ailleurs, je rappelle que nous avons déjà admis des souplesses en permettant aux départements et aux autres collectivités de participer au fonds national, qui, je le redis, s'élève à 7 milliards d'euros, avec plus de 6 milliards d'euros de participation de l'État et 500 millions d'euros des régions. Le Gouvernement encourage les communes, les EPCI et même les départements à participer à ce fonds national. Cette participation est évidemment très intéressante, parce qu'elle permet de coordonner nos forces. Je rappelle par ailleurs qu'à titre dérogatoire les collectivités qui participent à ce fonds national ...

Même si nous avons compris que le plan du Gouvernement était toujours en construction, la gravité de la situation et des enjeux impose de répondre rapidement à certaines questions clés. Celle des masques est essentielle, d'abord parce que la plupart des Français veulent en porter pour protéger les autres, mais aussi pour l'impact psychologique de leur port. Comme l'a rappelé notre collègue Jean-François Rapin, on vit une épidémie et le masque conforte les gestes barrières. Un géant français de la vente en ligne met en vente, avec votre accord, 60 millions de masques chirurgicaux pour les entreprises, alors que vous n'avez toujours pas répondu clairement aux pharmaciens, dont c'est pourtant le métier, qui vous interpellent pour savoir s'ils peuvent ou non vendre, à prix coûtant, des masques en tissu ou chirurgicaux, comme celui-ci. Pour les masques « grand public » promis par le Président, comment va s'effectuer cette distribution ? Si ce sont les collectivités qui en sont chargées, il faut leur dire comment se signaler,

auront-elles rapidement des consignes claires ? À trois semaines du déconfinement progressif, je relaye des questions simples de mes collègues : qui ? quand ? combien ? comment ? Si les collectivités s'en sont mieux sorties que l'État jusqu'à maintenant, notamment dans leur stratégie d'approvisionnement en masques chirurgicaux ou alternatifs, elles ont dès aujourd'hui besoin d'informations claires pour préparer cette

que les maires sont un maillon essentiel dans les territoires, car ils ont vocation à participer à cet effort collectif de protection de la population. La parole est

en ce début d'année, et qui va s'aggraver brutalement avec les pertes d'emploi, le chômage partiel et la disparition de l'entreprise. Beaucoup trop de nos concitoyens sont laissés sur le bas-côté nos étudiants, nos intérimaires, nos retraités, mais aussi les acteurs culturels, les organismes de solidarité- la liste est longue ... Le financement, essentiellement par le déficit et la dette, ne fait que renvoyer la charge à demain en la lissant. Il est urgent que les plus aisés, fortement avantagés depuis le début de ce quinquennat, prennent leur part à l'effort national. Alors même que la crise oblige à requestionner les paradigmes libéraux, le dogmatisme conduit le Gouvernement à préférer l'appel aux dons à la justice fiscale, le marché à la planification, l'incitation à la régulation. Ce PLFR ne permet pas, aujourd'hui, de définir de grandes orientations par rapport à l'après, notamment sur les politiques écologiques et environnementales, qui doivent pourtant constituer une réponse aux causes de cette épidémie. Il nous faut renforcer nos services publics sanitaires, mais pas seulement, notre souveraineté sanitaire et alimentaire, mais pas seulement. Il nous faut inventer un nouveau modèle de mondialisation ; notre pays a besoin d'un nouveau modèle économique, social, écologique. Cela se prépare dès maintenant, avec le Parlement, bien sûr, et en particulier avec cette assemblée. N'ayez pas peur du débat démocratique, car il est seul à permettre de trouver les réponses innovantes et partagées à une situation jusque-là inconnue ! N'ayez pas peur du débat sur la sécurité sociale, qui doit plus que jamais être préservée ! Mettez en discussion un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, même si rien ne vous y oblige.

que les bénéficiaires des APL recevront 100 euros par enfant. Ce sont 4 millions de ménages, monsieur le sénateur, qui seront concernés par ces aides. Le PLFR vise aussi à soutenir nos PME, nos TPE et nos entreprises en grande difficulté, notamment grâce au fonds de solidarité, qui passe de 1 milliard à 6 milliards d'euros, et au fonds de développement économique et social, qui passe à 1 milliard d'euros pour aider les PME et les TPE françaises. Enfin, un ensemble de dispositions auront pour objet d'aider toutes nos entreprises en difficulté

messieurs les ministres, mes chers collègues, nous vivons depuis quelques semaines avec une unique consigne : « Restez chez vous ! » Or arrive le moment où il va falloir redémarrer une vie sociale et professionnelle, au sens propre du terme « nous mettre en route », reprendre une mobilité. La question des mobilités a été au coeur de nos récents débats, ceux d'avant. Pour des raisons environnementales impérieuses, nous avions tous pris la mesure de l'enjeu des mobilités collectives. L'image des transports publics venait d'être mise à mal par les mouvements sociaux et l'impression d'une perte de qualité du service. Il fallait alors déjà regagner le coeur des usagers. À cela va désormais s'ajouter la peur pour sa santé, car la crise que nous traversons va poser d'énormes problèmes sanitaires dans les transports publics : difficile d'y respecter la règle de distanciation sociale, difficile d'éviter tout contact ; il faut pourtant restaurer la confiance et éviter à tout prix le retour en force du « tout-voiture individuelle ». Alors comment va s'organiser la gouvernance sanitaire des transports publics ? Qui va prendre les décisions ? Y aura-t-il une doctrine nationale ou cela relèvera-t-il de chaque autorité organisatrice de transport ? Quelles seront les mesures sanitaires ? Allez-vous rendre obligatoire le port des masques ? Où ? Lesquels ? Et si oui, qui les fournira ? Pourquoi pas également le port des gants ? Et sinon, comment est prévue la mise à disposition de gel Quelles modifications sont envisagées pour les procédures de nettoyage et avec quelles garanties pour l'usager ? Lors de son audition, M. Farandou nous expliquait que, en respectant la règle d'un mètre entre deux passagers, certains trains perdraient jusqu'à 80 % de leur taux de remplissage. Comment éviter l'asphyxie dans les transports urbains ?

Avant toute chose, je voudrais vous rappeler les mesures qui s'appliquent d'ores et déjà dans les transports publics, puisque nous avons édicté voilà maintenant plus d'un mois un décret qui porte obligation aux opérateurs de désinfecter tous les véhicules de transport au moins une fois par jour, qui interdit la vente des billets à bord, par exemple, ou encore qui impose d'équiper en masques certains opérateurs de transport particulièrement exposés. Ces mesures ont été adaptées en liaison avec les opérateurs, les autorités organisatrices et les organisations syndicales du secteur des transports.

les outils de protection sanitaire, vous avez cité le masque et la distanciation sociale. Ces mesures seront clarifiées et feront partie intégrante du plan. Mais nous travaillons aussi à l'amélioration drastique des procédures de nettoyage et de désinfection, à la régulation de l'emport maximal de personnels et de passagers dans les trains, vous l'avez cité, ou encore au lissage des heures de pointe, ce qui sera particulièrement précieux dans les métropoles à très forte densité de trafic. Toutes ces mesures seront connues et annoncées par le Premier ministre. Soyez assurée, madame la sénatrice, que nous mettons tout en oeuvre de manière que les passagers utilisent les transports dans de bonnes conditions, notamment sanitaires.

que, en gestion, nous pouvons faire face à des besoins en trésorerie ou en crédits de quelques millions d'euros, voire de quelques dizaines de millions d'euros, ne serait-ce que par la mobilisation de la réserve de précaution. nous veillons à ce que l'AEFE et ses établissements ne rencontrent pas de difficultés de trésorerie. Nous savons que la trésorerie de l'agence lui permet de faire face ; à ce jour,

Au mois de janvier dernier, l'Observatoire national de la précarité énergétique évaluait à près de 7 millions le nombre de personnes en situation de précarité énergétique en 2019 ; elles étaient ainsi 230 000 de plus

de celle en cours d'acheminement. Cette revalorisation offrirait un soutien aux ménages en situation de précarité énergétique pour le paiement de leurs factures d'énergie, dans la mesure où ils ne peuvent bénéficier du mécanisme de report de paiement, réservé aux microentreprises. Il y a bien d'autres raisons de soutenir cette revalorisation du chèque énergie,

un avis défavorable sur les trois amendements. Les dispositions et les engagements pris par le Gouvernement répondent aux problématiques exposées. La filière équestre sera accompagnée comme il se doit.

se sont engagés à financer. Je sais que Gérald Darmanin s'est engagé à transmettre au rapporteur général, ainsi qu'à tous les parlementaires qui le souhaiteraient, le projet de texte réglementaire qui encadrera ce dispositif. Je ne peux dire plus pour garantir que les engagements du Gouvernement seront tenus.

Une nouvelle fois, il faut faire le tri entre les annonces médiatiques du Gouvernement et ses actes. Le 7 avril dernier, Jean-Michel Blanquer annonçait la création de 1 248 postes d'enseignant dans le premier degré, conséquence du gel des fermetures de classes en zones rurales. Dix jours plus tard est déposé un projet de loi de finances rectificative comportant des mesures d'urgence. Surprise : la quasi-totalité des crédits ouverts concernent les aides aux entreprises et rien n'est prévu pour l'éducation nationale. Quand celle-ci deviendra-t-elle une urgence ? Cet été, quand les parents auront fait leurs choix d'inscription de leurs Quoi qu'il en soit, ces 1 248 postes sont essentiels, bien qu'insuffisants au regard des besoins, notamment dans les académies regroupant de nombreuses zones d'éducation prioritaire, qui restent les parents pauvres de ces nouvelles créations de postes. Ils sont essentiels à deux titres : d'abord, si ces postes ne sont pas créés, comment assurer le maintien des classes promis à la fin de mars, sauf à affaiblir encore le taux d'encadrement des élèves français

de 55 dans l'enseignement agricole. Comme l'a lui-même dit Emmanuel Macron le 13 mars dernier, les dernières semaines ont creusé encore un peu plus les inégalités sociales entre les élèves. Les prochains mois devront être marqués par un réinvestissement massif et la mise en place de dispositifs de soutien aux élèves les plus fragilisés. On ne peut se satisfaire de perdre de vue entre 600 000 et 960 000 élèves.

qui a salué nos fonctionnaires, personnels de santé, médecins, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers, secouristes, militaires, pompiers, pharmaciens, agriculteurs, enseignants, chauffeurs routiers, livreurs, électriciens, manutentionnaires, caissiers, caissières, éboueurs,

une prime de 500 à 1 500 euros nets pour les soignants engagés dans la lutte contre le Covid-19. C'est une somme très faible au regard de leurs sacrifices, qui n'ont pas commencé commencé avec cette crise. Depuis de longs mois en effet, le personnel soignant interpelle le Gouvernement sur la dégradation de ses conditions de travail, les fermetures de lits et les salaires au rabais. À titre d'exemple, selon une étude de l'OCDE publiée en 2017, le salaire d'un infirmier français s'élève à 0,9 fois le salaire moyen

M. Rémi Féraud. Cet amendement vise à compléter le plan d'urgence en créant un fonds de soutien doté de 2 milliards d'euros à destination du secteur touristique et hôtelier.

Nous avons entendu le Président de la République évoquer des annulations de charges plutôt que des reports. Gérald Darmanin lui-même a confirmé, le 15 avril, que l'État annulerait les charges pour les secteurs les plus touchés,

d'un amendement de ma collègue Claudine Lepage. Les salariés à domicile sont particulièrement impactés par la crise sanitaire. Certains ont vu leurs heures de travail drastiquement réduites, d'autres ont perdu leur emploi et, pour ceux qui continuent à travailler, le niveau de protection contre l'épidémie n'est pas satisfaisant. à cette crise sanitaire, la plupart de ces salariés se sont adaptés, modifiant les tâches qui leur incombaient, allant faire les courses et chercher les médicaments des personnes pour lesquelles ils travaillent, maintenant même parfois une présence physique ou téléphonique pour s'assurer de l'état de santé de celles-ci. On le voit, les salariés à domicile représentent souvent un maillon structurant et fondamental de la chaîne de prise en charge des malades et des personnes âgées à domicile. Les membres de notre groupe sont donc très attachés à ce que l'État fasse preuve de reconnaissance à l'égard de ces travailleurs. Un amendement en ce sens avait d'ailleurs été déposé par le groupe Socialistes et apparentés lors de l'examen du précédent PLFR à l'Assemblée nationale, mais le Gouvernement a choisi de s'en remettre à la bonne volonté des employeurs, ce qui nous paraît inacceptable. Cette solution déresponsabilise, une fois de plus, l'État.

Des réponses doivent être apportées d'urgence pour préserver ce pan essentiel de notre économie. Si le Gouvernement en a déjà mis certaines en oeuvre, les auteurs de cet amendement estiment

commune, la PAC, pour compenser dans la durée les pertes d'activité liées à la crise actuelle, dont les conséquences se feront certainement sentir sur plusieurs années. Ce futur fonds pourrait être cofinancé par l'Europe et les États membres, et permettrait également de préfigurer la part nationale d'un

par la cellule de veille, de contrôle et de suivi de crise de la commission des affaires économiques dédiée à l'agriculture. Elle renvoie par ailleurs à l'accord trouvé le 17 avril entre les vingt-sept ministres européens de l'agriculture pour activer au plus vite les instruments de régulation européens, de permettre la mise en oeuvre en urgence des mesures de soutien face à l'épidémie et, d'une manière plus générale, d'avoir une politique agricole commune qui soit plus protectrice de l'agriculture et de l'alimentation. D'autre part, l'ampleur de la crise devra nécessairement nous amener à nous interroger sur la question des reports de charges sociales actuellement mis en oeuvre. Dans certains secteurs particulièrement impactés, il faudra nécessairement transformer ces reports en exonérations totales, prises en charge par l'État. Ce fonds pourrait y contribuer dans un premier temps, pour les cas les plus urgents et critiques. En définitive, il assurera le bon fonctionnement de la chaîne agroalimentaire en apportant un soutien aux différents acteurs, et ce à tous les stades, de la production à la commercialisation en passant par la transformation, la logistique ou le stockage. Il s'agit bien évidemment d'assurer la bonne continuité de l'activité de l'ensemble d'une chaîne indispensable à la vie de notre pays et de préserver la diversité de l'agriculture française.

Si le Gouvernement a fait des annonces, rien n'est encore budgété. Or on sait qu'une annonce sans budget n'est que lettre morte. L'objet de cet amendement est donc de budgéter une prime de 1 000 euros destinée à l'ensemble des personnels des Ehpad afin de reconnaître leur travail, les difficiles conditions

des établissements accueillant des personnes handicapées. En raison de la multiplicité et de la diversité des employeurs dans cette filière- collectivités territoriales, secteur associatif, parfois acteurs privés

d'une attention particulière de la part des pouvoirs publics. C'est notamment le cas des productions saisonnières dont une part très importante du chiffre d'affaires est réalisée entre les mois de mars et de juin. Cette forte saisonnalité, conjuguée à la fermeture des points de vente habituels, plonge certaines filières dans une crise profonde, qui met en question leur pérennité même. pensent particulièrement aux filières ovine et caprine, qui bénéficient habituellement d'importants débouchés lors des périodes de fêtes religieuses des mois de mars et d'avril : agneaux, chevreaux et veaux sont alors particulièrement consommés. Ces animaux ne peuvent évidemment pas être stockés et doivent être vendus à ces périodes précises pour que les éleveurs puissent bénéficier de débouchés importants et de prix rémunérateurs. La filière gras est également fortement impactée avec la fermeture de la majorité des points de vente et le changement des habitudes de consommation, qui, en période de crise et dans le contexte anxiogène que nous connaissons, n'encouragent pas l'achat de ce type de produits, davantage considérés comme « festifs ». Il faut rappeler que cette filière a déjà été fortement touchée par plusieurs crises successives ces dernières années, liées à l'épizootie aviaire. Elle est aujourd'hui au bord de la rupture et il ne faudrait pas que cette nouvelle crise engendre sa disparition. Les auteurs de cet amendement estiment donc que, parallèlement aux mesures de soutien d'ordre général prises en faveur de notre agriculture, un effort financier spécifique doit être consacré en urgence aux productions saisonnières. C'est l'objet du présent amendement, qui prévoit la création d'un fonds de soutien exceptionnel doté de 400 millions d'euros.

concurrence de la dotation de 300 millions d'euros du nouveau programme ainsi créé, les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l'action n° 01 du programme 358, « Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire ». Quel

Le présent amendement vise à créer un fonds de soutien, doté de 300 millions d'euros, en faveur des associations de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, dans le cadre des mesures d'urgence

et au lien social. Chacun a pu voir aussi qu'une chaîne qui devait fermer en août, France 4, a permis à tous les enfants, notamment dans les zones non reliées à internet, d'avoir accès à des programmes éducatifs. Radio France,

Le présent amendement vise à créer un fonds permettant de couvrir une partie des pertes d'exploitation constatées, non prises en charge par les assurances, dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie, dans le cadre des mesures d'urgence prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19. La crise a entraîné la fermeture administrative des établissements de la restauration et de l'hôtellerie depuis le 14 mars, sans qu'aucun horizon de réouverture ne se dégage à ce stade, selon les premières informations communiquées par le Premier ministre lors de la conférence de presse sur les pistes d'organisation de la sortie du confinement Les mesures proposées par le Gouvernement ne sont clairement pas à la hauteur des enjeux pour certains secteurs, en particulier celui de la restauration et de l'hôtellerie. Les 1 500 euros d'aide au titre du fonds de soutien, par exemple, sont sans commune mesure avec les pertes de plusieurs dizaines de milliers d'euros par établissement subies ces dernières semaines. Dans l'immédiat, et compte tenu de l'urgence qu'il y a à prendre en compte la situation des entreprises de ce secteur en très grande difficulté, il est proposé de créer un fonds exceptionnel de compensation des pertes d'exploitation pour les métiers de la restauration et de l'hôtellerie. Quel avons déjà parlé des mesures qui permettent d'aider ce secteur. Avis défavorable.

Cet amendement vise à instaurer une mesure d'urgence sociale exceptionnelle en faveur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires, le Cnous, pour lui permettre de renforcer ses efforts en matière d'accompagnement des étudiants les plus en difficulté, en situation précaire ou isolés, dans le cadre de l'épidémie de l'épidémie de Covid-19. Cette mesure exceptionnelle permettrait avant tout au Cnous de suspendre purement et simplement l'appel des redevances jusqu'à la fin de l'année universitaire. En effet, si la décision du Cnous d'exonérer de loyers les étudiants qui ont pu regagner leur foyer familial est à saluer, nous pensons à ceux qui n'ont pu rentrer chez eux : les étudiants étrangers, isolés, en rupture familiale, dont la situation est souvent le plus précaire. Notre objectif est de permettre à tous les étudiants de finir leur année dans les meilleures conditions possible et de passer leurs examens ou concours, dont certains seront reportés et dont les modalités n'ont pas encore été définies.

doté de près de 50 millions d'euros en loi de finances initiale, pourront aussi être mobilisés. Nous avons mis en place un certain nombre d'actions, en matière d'accès à la prime d'activité, de suspension de loyers, d'accompagnement des étudiants les plus fragiles, qui nous paraissent répondre à votre objectif sans qu'il soit nécessaire de modifier la première loi de finances rectificative.

Ces latitudes sont mobilisées notamment pour répondre à la crise ; les moyens utilisés pour affronter la situation ne sont donc pas seulement ceux que l'on trouve dans les PLFR. C'est ce qui m'amène régulièrement à dire que ce que nous faisons par ailleurs à l'aide de crédits déjà votés et dans le cadre de dispositifs de droit commun suffit, si l'on peut dire, à répondre aux problématiques abordées par le biais d'amendements de crédits comme celui-ci.

a souhaité que les enfants puissent partir très largement en colonies de vacances ; encore faut-il que les organismes soient en mesure de les accueillir.

La question vous est posée de savoir s'ils devront payer un loyer ou s'ils en seront exonérés. C'est quand même une vraie question, à laquelle je trouve que vous devriez apporter une réponse

l'hôtellerie et de la restauration, qui sont dans une situation catastrophique, puisque plus de la moitié des établissements sont menacés dans leur existence même. Je vois que l'on s'apprête maintenant à répondre, concernant le tourisme social et les vacances des enfants

La protection de nos concitoyens les plus vulnérables est la première des exigences, comme l'a rappelé le Président de la République lors de son allocution du 13 avril dernier. Un jeune sur cinq vit actuellement sous le seuil de pauvreté et une grande partie des personnes sans domicile fixe ont moins de 25 ans.

et non bénéficiaires du RSA une aide exceptionnelle de 150 euros par mois de confinement. Cette aide exceptionnelle serait versée aux 1 220 000 jeunes de 18 à 25 ans vivant sous le seuil de pauvreté, afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins essentiels durant cette période de confinement. Je vous remercie,

je souhaite souligner que la prime d'activité ouverte aux jeunes actifs ou aux étudiants justifiant d'un revenu d'activité minimum constitue un premier socle d'aide. De la même manière, il existe une prime de précarité à laquelle les jeunes éligibles au RSA pourront prétendre, ainsi que les jeunes cohabitant avec leurs parents lorsqu'ils sont éligibles aux allocations logement. Pour les jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance (ASE), nous activons le dispositif « zéro sortie sèche de l'ASE », qui est intégré dans la stratégie de lutte contre la pauvreté et fait l'objet de contractualisations avec les départements. Nous avons également mis en place un programme spécifique d'aide alimentaire,

d'affaires entre le 15 mars et le 1 juin. Les conséquences de la crise actuelle sont donc très importantes pour elle. Or, si le Gouvernement a consenti à rouvrir les lieux de vente comme les jardineries ou les pépinières pour la commercialisation de semences et de plants potagers, il refuse toujours de le faire pour la vente de fleurs et d'arbustes. La filière chiffre ainsi les pertes potentielles dues à la crise entre 600 millions et 800 millions d'euros. Les auteurs de cet amendement souhaitent donc apporter une aide exceptionnelle à cette filière qui, à la différence d'autres secteurs, ne retrouvera pas ses stocks à la sortie du confinement. En effet, les plantes d'ornement sont vouées à la destruction si elles ne sont pas vendues dans les périodes où elles arrivent à maturité. Il est proposé, dans un premier temps, de doter ce fonds de 150 millions d'euros et de flécher ces aides sur les situations d'urgence, à savoir sur les entreprises dont la perte d'activité et de revenus subie remettrait en cause la survie. Quel

Soit nous défendons la continuité des services publics à l'étranger, dont on peut apprécier l'utilité en cette période de crise, et nous votons les crédits nécessaires à leur survie, soit nous procédons au démantèlement de l'AEFE-

un fonds spécifique destiné à aider les structures de droit étranger stratégiques pour les intérêts français et les Français de l'étranger. L'amendement

De plus, les événements culturels au titre desquels elles sont subventionnées ne peuvent plus se tenir. Les bibliothèques sont fermées. Les personnels, souvent vacataires, y compris les professeurs, se retrouvent sans emploi. Les petites Alliances françaises, en particulier, peinent à survivre et risquent de devoir mettre la clé sous la porte. Certaines quittent désormais des locaux dont elle ne peut plus payer le loyer.

où il n'y a pas d'allocations chômage pour garantir les postes des personnels et la pérennité du réseau. Ce sont en effet des centaines d'enseignants de français langue étrangère qui risquent de se retrouver sans emploi. On peut craindre que l'apprentissage du français ne représente pas forcément, demain, un poste de dépense prioritaire pour les familles et les entreprises. Certaines Alliances enregistrent d'ores et déjà une perte de près de 70 % de leurs étudiants. Elles réalisent en France une grosse partie de leur chiffre d'affaires durant la période estivale, en recevant des étudiants du monde entier en séjour linguistique. Avec la fermeture des frontières, on peut craindre une nouvelle perte de recettes massive. Au-delà de l'enseignement de proximité de la langue française qu'elles dispensent, les Alliances françaises à l'étranger

Ce fonds serait doté de 75 millions d'euros. Les conditions de réouverture des écoles, le 11 mai, suscitent encore beaucoup de questions, mais elles commencent à être explicitées. Le ministre de l'éducation nationale a

que vous indiquiez à chaque étape qu'il faudrait faire différemment. Nous sommes au Parlement, nous examinons un projet de loi de finances rectificative et sommes en train d'identifier les secteurs dans lesquels il faudrait intervenir. Vous n'êtes pas chef du Gouvernement, ou pas encore,

toutes les dispositions sur la présence économique française à l'étranger ne sont pas traitées, alors qu'il y a urgence ! Il ne faudra pas se réveiller dans deux ou trois mois, quand on n'aura plus de chambres de commerce.

de vote. Je vais aller dans le sens du rapporteur général. Cette discussion est intéressante. Pour ma part, je pense que la stratégie sanitaire de lutte contre l'épidémie est totalement imbriquée dans la stratégie économique, et c'est parce que l'on a une mauvaise stratégie sanitaire que l'on sera l'un des pays européens qui restera confiné le plus longtemps. La première vague de déconfinement

chroniques. Si nous avions une stratégie de tests systématiques et de masques généralisés, nous pourrions rouvrir plus tôt. Telle est la réalité. Eh oui ! Si nous en restons là, le coût économique sera énorme : nous n'aurons pas tué le virus-

Pour pouvoir dire aux Français qu'ils peuvent ressortir en toute sécurité, il faut soit qu'ils aient tous été vaccinés- on évoque un horizon d'au moins un an -, soit que 60 % à 70 % de la population aient été en contact avec le virus ; c'est la loi de Charles Nicolle, bien connue des épidémiologistes. Les études dont nous disposons aujourd'hui indiquent que 3 % à 10 % des Français ont été en contact avec le virus. Si je retiens le chiffre du Gouvernement qui est le plus favorable, cela doit être de l'ordre de 10 % ; c'est ce qui a été communiqué ces jours-ci. Si nous devons attendre de passer de 10

il n'existe pas de vaccin, le taux de contamination est très faible et notre économie ne survivra pas à trois ou quatre mois de confinement supplémentaires. Il faut en tirer les conséquences courageusement et dire la vérité aux Français.

par la crise. Au-delà des problématiques liées à la main-d'oeuvre, à la saisonnalité de certaines productions et à la commercialisation des produits du fait de la fermeture des lieux de vente, il existe également un manque à gagner important avec l'arrêt total des activités liées à l'agritourisme. Le tourisme rural représente un tiers de la fréquentation touristique en France, et l'agritourisme y prend une place croissante depuis quelques années. En effet, ce secteur est en plein essor du fait de l'intérêt croissant des Français pour redécouvrir le savoir-faire agricole d'un territoire, mais également des exploitants agricoles, afin de partager leurs métiers et leurs passions. Ainsi, outre qu'il crée de l'activité et du lien social en zone rurale, l'agritourisme offre une diversification importante, et souhaitable, du revenu des agriculteurs.

Monsieur le secrétaire d'État, à l'Assemblée nationale, vous avez mentionné l'utilisation de la soulte pour aider les besoins complémentaires. Mais si elle devait être utilisée pour l'octroi de bourses exceptionnelles, elle ne serait certainement pas suffisante. nous sommes aujourd'hui dans l'incapacité de connaître l'ampleur de l'impact de la crise économique sur les familles et leurs capacités à y faire face. Les commissions locales de bourses qui se tiennent ou vont se tenir bientôt devraient nous y aider, mais nous sommes tous dans l'estimation au doigt mouillé, comme le dit Claude Raynal, des demandes à venir. Cependant, s'il n'y a pas de consensus sur les montants, il y en a un sur la nécessité absolue d'anticiper une demande supérieure à la normale. Après

dans ce PLFR, quand le sera-t-il ? On imagine mal des annonces sans suite, surtout quand elles sont publiées sous le sceau du ministère. En tout cas, sachez que nous soutenons le ministère de l'Europe et des affaires étrangères ; cette proposition l'atteste.

ce sujet. Un rapport annuel de la Fédération française de l'assurance indique que les stocks constituent 1,4 % de la provision mathématique des fonds.